Mes chers collègues, par lettre en date du 3 août, le Gouvernement sollicite du Sénat l'inscription de la proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce à l'ordre du jour de la séance du mercredi 5 octobre 2022 après-midi. Y a-t-il des observations ? observations ? ... Il en est ainsi décidé. Nous pourrions inscrire l'examen de ce texte en dernier point de l'ordre du jour de l'après-midi et prévoir une discussion générale de trente minutes. La commission des lois se réunirait pour le rapport et le texte le mercredi 28 septembre au matin. Le délai limite de dépôt d'amendements de séance sur ce texte serait fixé au lundi 3 octobre, à douze heures. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale n'ayant pas tout à fait achevé l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative, nous sommes tenus d'attendre. Je vais donc suspendre la séance, qui sera reprise

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission n°

sur ces points. Enfin, la question d'un nouveau dépôt se pose, notamment pour arrêter les comptes en comptabilité générale et pour les affecter au bilan de l'État, en vue de faciliter leur certification par la Cour des comptes. À ce stade, l'opportunité juridique et comptable d'un nouveau dépôt fait l'objet

concrètement consacrée par nos décisions ; deuxièmement, le soutien aux collectivités locales, acteurs de proximité reconnus et appréciés dans la mise en oeuvre des services quotidiens pour nos concitoyens ; troisièmement, l'arrêt de la dégradation de nos comptes publics. publics. La valeur travail est reconnue et soutenue, dans un contexte de retour de l'inflation qui pèse à la fois sur les ménages et, malheureusement, sur les entreprises, au travers d'une pénurie de main-d'oeuvre.

du plafond applicable pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Elle a ensuite étendu jusqu'au 31 décembre 2025 la possibilité offerte aux salariés, avec l'accord de l'employeur, de convertir en majoration de salaire tout ou partie

nous sommes accordés sur la nécessité d'allouer une aide exceptionnelle de rentrée à tous les bénéficiaires de la prime d'activité, au même titre que les allocataires des minima sociaux.

à destination des associations d'aide alimentaire, soumises à d'importantes difficultés d'approvisionnement, pour permettre à tous les Français de se nourrir chaque jour. Ensuite, le Sénat s'est engagé à garantir aux collectivités territoriales les moyens de leur action.

au titre de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation. Nous avons renforcé le « filet de sécurité » introduit par l'Assemblée nationale, nous inscrivant dans les pas

Bruno Le Maire l'a souligné ce matin, c'est une triple victoire : une victoire pour les Français, qui pourront mieux faire face à l'augmentation des prix ; une victoire de la politique du compromis ; enfin, une victoire pour les finances publiques, qui ont été tenues. Ce PLFR a été examiné par le Parlement après la publication des derniers résultats de l'économie française. Avec un chiffre de croissance de 0,5 % pour le deuxième trimestre 2022, la France obtient l'un des meilleurs résultats de la zone euro.

Vous le savez, nous sommes dans le pic inflationniste. Cette inflation restera probablement à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2022. Nous avons cependant de bonnes raisons d'espérer une baisse de celle-ci dans le courant de 2023 ; j'y reviendrai plus tard. Il s'agit donc d'un cap à passer. Et avec ce paquet pouvoir d'achat, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour accompagner nos compatriotes dans cette période. Grâce à l'accord trouvé en CMP, nous maintiendrons le « bouclier énergie » jusqu'à la fin de l'année 2022, avec le gel du prix du gaz, d'une part, et le plafonnement de la hausse du prix de l'électricité à 4 %, d'autre part, alors que, je le rappelle, cette dernière hausse aurait été de 45 % sans notre intervention. Ce bouclier énergie nous permet d'avoir le taux d'inflation le plus faible de la zone euro. En effet, et vous le savez déjà, l'inflation est tirée à 50 % par le seul prix de l'énergie. Je veux vous redire, au nom du Gouvernement, que nous continuerons également à nous battre au niveau européen pour dissocier définitivement le prix de l'électricité décarbonée du prix du gaz. Nous avons par ailleurs trouvé un compromis sur le fioul, M. le rapporteur général l'a rappelé. Il comprend l'adoption d'une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui utilisent ce combustible pour se chauffer. Nous proposons d'associer les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat au ciblage des ménages qui pourront bénéficier de cette aide supplémentaire. Jusqu'à 3 millions de ménages français sont concernés. Nous allons faire passer la ristourne sur les carburants à 30 centimes d'euros en septembre, à 30 centimes en octobre, à 10 centimes en novembre et à 10 centimes en décembre. Pour les Français qui travaillent, d'autres dispositifs seront mis en place. Nous avons voté le doublement du plafond d'exonération de la « prime carburant » versée par les employeurs, de 200 à 400 à 400 euros. Nous allons aussi permettre son cumul avec la prise en charge de l'abonnement transport collectif. Nous avions, par ailleurs, déjà revalorisé de 10 % le barème kilométrique de l'impôt sur le revenu en 2022. Nous sommes prêts à le revaloriser de nouveau en 2023. Ce PLFR vise également à rendre du pouvoir d'achat aux Français par la valorisation de leur travail. Je sais combien vous y êtes sensibles. La mesure de monétisation des RTT permettra aux salariés qui le souhaitent de travailler plus afin d'augmenter leur rémunération, dans des conditions fiscales avantageuses. Concernant la défiscalisation des heures supplémentaires, le relèvement du plafond d'exonération fiscale de 5 000 euros à 7 500 euros est une bonne chose ; grâce au Sénat, cette mesure devient pérenne. Enfin, grâce aux discussions entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les entreprises de 20 à 250 salariés verront leurs charges sociales patronales réduites de 50 centimes par heure supplémentaire travaillée. Je veux remercier le président Retailleau, qui a soutenu ce projet. aujourd'hui devant l'assemblée des collectivités locales. Je sais que l'inflation et que les revalorisations engagées peuvent susciter des inquiétudes. Sur l'initiative de Mme Christine Pires Beaune, les députés ont adopté à une large majorité le dispositif suivant. voté 180 millions d'euros de crédits ciblés s'adressant aux plus de 6 000 communes qui sont en difficulté, parce qu'elles peinent à faire face à la hausse du prix de l'énergie et à celle du point d'indice. Les collectivités d'outre-mer sont particulièrement concernées, et je sais que vous y êtes sensibles. ont voté 120 millions d'euros pour compenser la hausse du RSA au niveau des départements. Au Sénat, un nouveau compromis a été trouvé grâce au rapporteur général Jean-François Husson. Je veux également saluer le travail du président François Patriat et du président Hervé Marseille sur ce sujet. Ce sont ainsi près de 22 000 collectivités qui bénéficieront finalement de ce filet de sécurité. Durant les débats, l'idée de taxer les surprofits est arrivée. Comme à l'Assemblée nationale, cette idée a été rejetée par la Haute Assemblée, et je tiens à saluer la sagesse du Sénat. Bruno Le Maire l'a rappelé, alors que nos compatriotes souffrent de la vie chère, nous partageons tous l'idée selon laquelle chacun doit porter une part du fardeau de l'inflation : l'État, bien entendu, qui le fait déjà ; les ménages, qui y sont contraints avec l'augmentation des prix alimentaires et des prix des carburants ; et, bien sûr, les entreprises. Je ne conteste pas ce raisonnement. Toutefois, l'immense majorité des entreprises souffrent de l'inflation. Elles sont de toutes les tailles- grandes entreprises, ETI, PME, TPE -et opèrent dans tous les secteurs. Les entreprises du bâtiment et des transports sont lésées par l'augmentation du prix des matières premières. Les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, de la distribution sont lourdement pénalisées par le manque de main-d'oeuvre. Nombre d'entreprises participent en réalité déjà à la lutte contre l'inflation en augmentant les salaires.

En revanche, quelques entreprises font des bénéfices importants, c'est vrai. Elles doivent participer à l'effort collectif, à l'image de la remise de 20 centimes à la pompe pour TotalEnergies, de la baisse du prix des conteneurs pour CMA-CGM ou du chèque énergie pour Engie. Cette approche est tout simplement plus juste, plus efficace et plus conforme à vos aspirations pour nos territoires. Elle est plus juste, car elle ne pénalise pas des entreprises qui ont besoin d'investir pour leur avenir et la pérennité de l'emploi. plus efficace, car l'argent va directement dans la poche de nos compatriotes : 20 centimes de remise à la pompe, cela amène le litre de carburant à 1,50 euro, une fois cette remise combinée avec la ristourne que vous avez votée. plus conforme à vos aspirations, car elle va dans le sens de la baisse des impôts, qui est notre ligne et qui favorise l'attractivité de notre territoire, de tous nos territoires. Du point de vue des finances publiques, nous observons que, en baissant les impôts, nous obtenons plus de recettes fiscales. Je pense, par exemple, à la baisse de notre taux d'impôt sur les sociétés, qui s'est accompagnée accompagnée d'une augmentation de son produit entre 2017 et 2022. En libérant de la capacité à investir, nous avons permis à nos entreprises de créer plus de richesses, c'est un fait. Enfin, ce PLFR acte la suppression de la contribution sur l'audiovisuel public, qui rendra 138 euros de pouvoir d'achat aux ménages. Cette décision est conforme à notre politique de baisse des impôts, à laquelle les sénateurs sont attachés, me semble-t-il. L'Assemblée nationale a travaillé à un dispositif de financement durable de l'audiovisuel public, gage de son indépendance. Tâchons de poursuivre ce dialogue constructif. Pour conclure, comme je l'ai dit au début de mon propos, ce paquet pouvoir d'achat arrive au bon moment, puisqu'il aidera nos compatriotes à passer ce cap difficile. Je reste confiant dans notre capacité collective, en France et en Europe, à ramener l'inflation à un taux raisonnable dans le courant de l'année 2023. Nous pouvons compter sur les mesures prises par la Banque centrale européenne (BCE) en matière de politique monétaire. Surtout, nous agissons chaque jour par les mesures que nous prenons en matière d'énergie et de diversification de nos approvisionnements. En mai dernier, les Français ont réélu Emmanuel Macron Président de la République. Fin juin, ils ont également voulu marquer une autre volonté, celle de voir les différentes forces politiques du pays dialoguer et trouver des compromis

commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous allons maintenant adopter les termes a été débattu dans un calendrier strict, entre deux bornes : d'une part, la reprise des travaux parlementaires après l'élection de l'Assemblée nationale ; d'autre part, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour aider les Français et les acteurs économiques à surmonter les effets de l'inflation qui nous pressent.

et je crois que nous sommes nombreux à souhaiter que, au terme de cette consolidation, nous sortions définitivement de la mauvaise habitude consistant à financer des dépenses de fonctionnement et de solidarité avec des emprunts.

l'augmentation des minima sociaux et du SMIC et, spécifiquement dans ce texte, l'aide exceptionnelle de rentrée et le soutien aux associations d'aide alimentaire. Deuxièmement, soutenir les revenus d'activité, ce qui se traduit, au-delà des revalorisations salariales, par la revalorisation des exonérations de titres-restaurants, par l'exonération fiscale améliorée de 50 % des heures supplémentaires et par la compensation partielle en monétaire en monétaire des RTT- l'équivalent pour les bénéficiaires de RTT de l'exonération des heures supplémentaires -, et cela pour une période de trois ans. En revanche, et je sais que cela a donné lieu à des interventions critiques, il n'a pas été prévu de mesures

Il ne fallait donc pas introduire trop de discriminations entre les collectivités et adopter des critères larges. C'est ce qui a été fait, et nous en sommes satisfaits, non pas seulement sous un angle politique et d'équité, mais aussi avec une préoccupation

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a deux cent trente-trois ans jour pour jour, le 4 août 1789, l'Assemblée constituante abolissait les privilèges, ce qui devrait prouver aux esprits chagrins que le Parlement peut voter des textes importants en plein été, et même en pleine nuit. C'est le cas aujourd'hui, toutes proportions gardées bien sûr, avec l'adoption du paquet pouvoir d'achat, qui vise à atténuer les violents effets de l'inflation sur nos concitoyens. Le sujet était aussi complexe que sensible. Je crois que nous sommes parvenus à un texte équilibré, qui comporte de nombreuses mesures concrètes, dont les Français mesureront vite les pleins effets. C'est ce qu'ils attendaient de nous. C'est que nous avons fait. En la matière, les remèdes miracles n'existent pas. Tout est question d'équilibre et de dosage : augmenter le pouvoir d'achat sans doper l'inflation ; hausser les rémunérations sans baisser la compétitivité ; et, surtout, ne pas creuser le déficit public. Il y a quelques années, quelques mois encore, les économistes débattaient dans le confort de leur chaire pour savoir si l'inflation appartenait à l'histoire ancienne. Par empirisme ou par dogmatisme, ils soutenaient qu'elle avait disparu de nos contrées, comme jadis la peste ou les tyrannies. C'était avant 2020. Puis il y a eu la pandémie, puis le confinement généralisé, puis la reprise économique dopée par un keynésianisme sous stéroïdes, puis un choc de demande sans augmentation d'offre, et, enfin, le grand retour de l'inflation. Et il y a eu surtout le retour de la guerre en Europe, la folie meurtrière du boucher du Kremlin, sa haine obsessionnelle de la démocratie et de la liberté. La donne a changé. Rien n'indique que les choses rentreront bientôt dans l'ordre. Le jusqu'au-boutisme de l'ex-colonel du KGB contre la résistance héroïque des Ukrainiens, les risques de famine qui pèsent sur l'Afrique par sa faute, les menaces de la Chine sur Taïwan, les populismes qui gangrènent l'Europe, sont autant de menaces qui imposent la plus grande vigilance. Ce monde inquiétant doit nous donner le courage et l'ambition de poursuivre nos efforts pour renforcer la souveraineté nationale et de mettre à profit ce budget rectificatif, le premier du quinquennat qui s'ouvre, pour lancer quelques réformes importantes. Ce fut le cas sur la question, très sensible au Sénat, des surcoûts liés à l'inflation et supportés par les collectivités et de leur compensation par l'État. Le point d'équilibre trouvé entre le Gouvernement et le Sénat prévoit une juste répartition du fardeau entre État et collectivités, tant sur les dépenses liées au RSA que sur celles qui dépendent du point d'indice. Ce budget revalorise également le travail, en activant plusieurs leviers fiscaux qui porteront rapidement leurs fruits. Je pense notamment à la défiscalisation des heures supplémentaires. Nous sommes nombreux ici à soutenir de longue date cette mesure. Dans la même logique, la possibilité donnée aux salariés de racheter leurs RTT doit permettre à ces derniers d'augmenter leur rémunération par leur travail, n'en déplaise à ceux qui hurlent à la « casse sociale » et à la fin des 35 heures, ces 35 heures qui ont précipité notre déclassement et qui préfiguraient l'incroyable allergie au travail qui s'abat depuis quelques mois sur tant de nos concitoyens. Si seulement une telle mesure pouvait nous permettre de rompre, pour de bon, avec l'illusion tenace selon laquelle le travail est un gâteau à partager à parts égales, ce texte serait un pas dans la direction du redressement national. Le Président de la République, à l'instar de l'un de ses prédécesseurs, nous a récemment rappelés à l'évidence : pour financer notre modèle social, garantir notre souveraineté économique et accélérer la transition écologique, il nous faudra travailler plus. Le Sénat est prêt à le soutenir pour oeuvrer dans ce sens. J'espère que nous serons au rendez-vous pour soutenir les mesures difficiles, mais nécessaires au rétablissement des finances publiques. Nous avons suivi le Gouvernement dans sa volonté de ne pas céder à la facilité des contributions exceptionnelles, taxes extraordinaires et autres innovations fiscales, qui s'inscriraient dans le droit fil de la pratique qui nous ronge depuis des années et que j'ai déjà dénoncée ici tout ce qui bouge, on le taxe ; tout ce qui bouge encore, on le réglemente ; tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. Pour désendetter l'État dans le pays champion du monde des prélèvements obligatoires, l'alternative entre baisser les dépenses et augmenter les taxes n'existe pas. Il faut baisser les dépenses Et comme l'inflation pousse les taux d'intérêt à la hausse, nous allons redécouvrir que s'endetter a un coût, que nous ne pouvons plus nous permettre sans renoncer à des priorités essentielles. Le « quoi qu'il en coûte » nous a permis de tenir bon et de surmonter la crise sanitaire, économique et sociale. Il était nécessaire. Mais il faut désormais remettre de l'ordre dans nos comptes, pour nous préparer aux défis qui s'annoncent. La parole

la CMP qui s'est réunie hier soir est parvenue à un très bon accord, sur un texte particulièrement important, qui vise la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Les débats ont été longs et intenses et ils ont permis, me semble-t-il, à tous les groupes de défendre leurs propositions pour soutenir les Français marqués par la hausse de l'inflation. Pour ce qui concerne le groupe Les Républicains, notre ligne a été très claire le soutien au pouvoir d'achat des ménages passe d'abord par la valeur du travail, et certainement pas des chèques temporaires financés par de la dette. Dans cet esprit, nous avons porté et fait adopter des mesures puissantes pour acter définitivement la fin des 35 heures, signe d'appauvrissement des Français et d'affaiblissement de notre économie. C'est le cas avec la pérennisation des heures supplémentaires défiscalisées, inscrites dans le texte de la CMP. C'est également le cas avec le rachat optionnel de RTT, rendu possible jusqu'à la fin de 2025- en espérant que cette mesure devienne pérenne. C'est un signe de responsabilisation et de liberté offerte aux salariés, cadres et non-cadres, qui permettra un complément de revenu important. Par ses votes, le Sénat a également envoyé des messages très forts aux collectivités, qui font face à un coût de l'énergie de plus en plus élevé et qui doivent subir la hausse du point d'indice de la fonction publique. La majorité sénatoriale est parvenue, avec le Gouvernement, à un accord ambitieux en séance. Cet accord a été confirmé en CMP, et je m'en félicite. Demain, plus de la moitié des communes françaises pourront bénéficier d'une dotation exceptionnelle pour tenir durant cette période compliquée. Je me réjouis également de l'adoption conforme, par nos deux chambres, de la compensation intégrale de la hausse du RSA pour les départements. Et nous n'avons pas oublié les régions, qui bénéficieront d'une compensation pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. Sur la proposition de notre rapporteur général, que je remercie du travail qu'il a réalisé et de sa pugnacité, nous avons complété plusieurs dispositifs initialement proposés. Je pense au soutien de 40 millions d'euros accordé aux banques alimentaires, ou encore aux renforts financiers fléchés vers les Mes chers collègues, après le vote de ces mesures d'urgence, il nous faudra préparer l'avenir. Nous ne pourrons pas collectivement nous satisfaire, dès qu'une crise survient, d'ouvrir les vannes de la dépense publique en créant des chèques et des ristournes. Agir efficacement pour le pouvoir d'achat, c'est, je l'ai dit, encourager le travail, combattre le chômage et lutter contre le déficit de la balance commerciale. C'est également mieux cibler les aides et nous obliger à les rendre temporaires. C'est, enfin, parvenir à un État plus agile, moins endetté et moins drogué à la dépense publique. Dans le texte de la CMP, et sur l'initiative du Sénat, nous avons obtenu deux mesures importantes à ce sujet. Tout d'abord, la création d'une carte Vitale biométrique, remède nécessaire aux milliards d'euros de fraude qui privent l'assurance maladie de recettes capitales. Ensuite, la suppression de 1 milliard d'euros- même si nous demandions 4,5 milliards d'euros -de crédits sollicités par le Gouvernement, mais non affectés à une dépense précise. C'est tout à la fois une mesure d'économie efficace et un signe de respect des assemblées parlementaires. Mes chers collègues, le second quinquennat du Président de la République ouvre de nouvelles perspectives pour la démocratie et pour le Sénat. En témoignent les très nombreuses dispositions issues de notre chambre qui seront prochainement promulguées et qui auront force de loi. Nous pouvons et nous devons nous en réjouir et continuer d'oeuvrer ensemble pour le redressement économique et financier de notre pays. Le groupe Les Républicains votera ce PLFR, fruit de l'accord trouvé hier en commission mixte

pour tenir compte des difficultés incontestables auxquelles font face les Françaises et les Français les plus modestes, pour tenir compte des troubles climatiques qui chaque jour saccagent notre biodiversité, déroutent nos agriculteurs, assèchent nos terres ou encore brûlent nos forêts, pour tenir compte des conséquences de la guerre en Europe menée par Poutine, pour suivre une stratégie énergétique sobre et d'avenir. Vous aviez cette possibilité, monsieur le ministre, avec ce PLFR. Vous aviez ce pouvoir. Vous aviez même, selon le groupe écologiste, ce devoir. Il y eut des rectifications et des mesures bienvenues, même si elles restent très inférieures à l'inflation. Ainsi, nous saluons une rectification, celle que la CMP a apportée en rétablissant l'aide exceptionnelle de rentrée pour les bénéficiaires des minima sociaux.

sont les plus malmenés par la crise : vous ne les aidez pas, pas assez ou trop peu ... Ils rencontrent des difficultés pour se loger, se nourrir et se soigner. Vous revalorisez les bourses, mais pas à la hauteur de l'inflation. (Crous) devront faire face à l'augmentation des prix. Les universités sont au bord de l'asphyxie, avec des moyens de plus en plus contraints et des difficultés structurelles importantes, et souvent des bâtiments énergivores. Étudier est un droit, pas un privilège. L'éducation, la jeunesse et l'enseignement supérieur sont des investissements nécessaires pour notre pays, avant d'être des dépenses. Ils devraient donc être valorisés.

cette mesure vient du Sénat -, ce qui aidera peut-être à maintenir dans le giron de la majorité les sénateurs centristes. Mais vous prévoyez aussi une réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités de 0,5 % par an, sur la période 2022-2027, dans le pacte de stabilité Alors, oui, vous avez rétropédalé dans une formule très claire du ministre Christophe Béchu, qui y voit « une modération des dépenses de fonctionnement, pour qu'elles augmentent en moyenne annuelle de 0,5 % de moins que leur tendance naturelle Cette phrase est très claire, mais je serai plus direct : cette modération est une baisse, et rien de plus. S'agissant de l'audiovisuel public, vous avez fait preuve de l'impréparation la plus totale, et le dispositif auquel on aboutit est instable. Je retiens la proposition de Mme la ministre Rima Abdul-Malak d'un débat national.

Ces deux mesures indispensables, mais, avouons-le, encore modestes, n'ont même pas été conservées en CMP. Que d'occasions manquées ! Votre modèle charge le déficit public de 20 milliards d'euros et ne prend rien aux profiteurs de crise qui bénéficient de dizaines de milliards d'euros non imposés. Nous ne comprenons pas que l'on se prive de la ressource de la taxation des superprofits à l'heure où nos services publics sont mis à mal. L'Union Centriste défendait ces mesures de bon sens que, sur les travées de la gauche et des écologistes, nous portons avec conviction et constance. J'entendais J'entendais parler ce matin de votre stratégie de dialogue et de compromis, comme si c'était une opportunité ... Le compromis est, hélas, à ce jour, assez clair et lisible : l'accord entre deux visions libérales, la vôtre, monsieur le ministre, et celle des Républicains, est scellé. Vous êtes revenus sur des fondamentaux, comme la question du temps de travail. Vous monétisez le temps libre au risque de la santé des salariés et vous excluez les partenaires sociaux. Vous avez choisi de subventionner les week-ends en SUV, ou, plutôt que de réserver les aides aux salariés qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller Pas d'investissement non plus dans les alternatives douces : c'est navrant ! Nos propositions demeurent, même si certains préfèrent ici nous chahuter plutôt que nous écouter. Or les scientifiques ont lancé, avant-hier encore, un nouvel appel face à la gravité des crises à venir. René Dumont, lui aussi, était moqué lorsqu'il annonçait, en 1974,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la séquence dédiée aux mesures de pouvoir d'achat se clôt ici, au Sénat, dans la confusion budgétaire et le déficit démocratique. Confusion budgétaire, car le Parlement a rejeté, pour la seconde fois de son histoire, la loi de règlement pour 2021. Ainsi, contrairement à ce que vient d'affirmer M. le ministre, lois de finances (LOLF), la prochaine loi de finances ne pourra être examinée sans un vote positif du Parlement sur les comptes de la Nation pour 2021. Les manipulations comptables du Gouvernement sont apparues au grand jour : il n'y a pas de « trésor de guerre », de surplus de recettes cachées. Pour preuve, le solde budgétaire n'est en excédent que de 2,6 milliards d'euros par rapport aux prévisions. Déficit démocratique, car, à l'issue du conclave de la CMP, la fumée blanche entérine le rapprochement du Gouvernement et de la droite sénatoriale, satisfaisant aussi le Rassemblement national et ses députés. Les débats parlementaires ont été préemptés par des accords préalables, des accords de couloir, au détriment de la transparence démocratique des débats dans l'hémicycle. Les surprofits indécents des multinationales ne serviront pas à financer en bout de elles qui, comme nos compatriotes, sont frappées de plein fouet par la spéculation et la course au profit. L'audiovisuel public et son indépendance constitutionnellement garantie sont maintenant menacés par la suppression de la redevance. Quand l'accord entre les droites passe, la justice fiscale et les services publics trépassent ! Pourtant, à l'issue de la séquence électorale, une partie du peuple n'a pas opté pour ce projet politique. Vous n'en tenez pas compte. Les deux lois sur le pouvoir d'achat comportent des invariants l'inflation augmente sur un an de 6,1 %, sans qu'aucune des mesures prises préserve intégralement le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ce sont 2 points de pouvoir d'achat perdus pour les allocataires des minima sociaux. Ce sont 2,5 points perdus en plus s'ils sont locataires, au profit des rentes privées. Au cours de ces débats, nous n'avons eu de cesse de vous proposer des mesures de substitution à même d'enrayer la spirale inflationniste. Parce que c'est un impôt insidieux sur les ménages modestes et les classes moyennes, nous continuons de porter le blocage des prix : à la pompe, sur les factures d'énergie, pour les loyers et les produits alimentaires de première nécessité. Le consensus des droites a évacué avec un certain mépris la question des salaires. En revanche, il s'est agi d'inventer toutes les mesures accessoires à la rémunération du travail, avec une constante aucune des contributions des entreprises n'est obligatoire. Alors, selon leur bon vouloir, elles pourront verser la prime Macron, doubler le montant de l'aide carburant pour leurs salariés ou augmenter de quelques centimes les tickets-restaurant. En somme, aucune obligation cela ne vous suffit pas ... Les travailleurs en sont quittes pour sacrifier leurs droits au repos, avec une remise en cause sans précédent des 35 heures par la monétisation de leurs RTT. Ce sont les salariés les plus précaires qui, faute de mieux, devront concéder sous la pression du patronat leurs jours de repos. Le rehaussement du plafond des heures supplémentaires est une autre entorse faite au code du travail. En somme, la morale libérale institue le « travailler plus », faute de gagner plus ! Ensuite, la droite sénatoriale, dans une forme de surenchère dramatique, oppose les allocataires des minima sociaux aux travailleurs pauvres. Ces relents créent un clivage nauséabond et factice entre les bons citoyens et ceux qui ne prendraient pas leur part à l'activité économique de la Nation. La négation de ce qu'est la réalité du « marché de l'emploi » est coupable. près de 15 millions de contrats de moins d'un mois ont été signés, qui représentent 64 % des embauches réalisées ! Dès lors, comment avez-vous osé proposer une réduction de quelques euros pour les allocataires du RSA ? Comment avez-vous osé exclure d'un chèque plus de 4 millions de foyers pauvres et 1,8 million d'étudiants, dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté ? La CMP est revenue sur cette disposition inique, sans pour autant garantir le montant de l'allocation versée. Enfin, le fameux « miracle républicain » destiné à soutenir nos collectivités territoriales n'a pas eu lieu. Ce simulacre d'accord trouvé sur la compensation de la revalorisation du point d'indice, de la hausse du RSA, de la hausse du prix de l'énergie et des denrées alimentaires est indigne de la chambre qui prétend représenter les collectivités territoriales. Alors que celles-ci sont déjà privées de leurs recettes fiscales. Vous portez là un nouveau coup à leur libre administration, par la non-compensation de décisions prises par l'État central. La conclusion de ces débats ne laisse que des perdants

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire réunie hier soir a abouti à un accord. Je tiens à féliciter les deux rapporteurs généraux pour leur travail efficace et constructif, dans un temps si contraint. Le groupe Union Centriste a abordé l'examen de ce premier projet de loi de finances rectificative de l'année 2022 avec une doctrine claire et cohérente : privilégier les mesures temporaires et ciblées, en conciliant justice sociale et réduction de la dette. Nous avons soumis à la discussion plusieurs propositions allant en ce sens. Des motifs de regrets demeurent à cet égard, et l'examen, dont la perspective est déjà proche, du projet de loi de finances pour 2023 sera pour nous l'occasion de revenir à la charge.

tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs et à utiliser les fonds pour soutenir les plus vulnérables en ces temps difficiles ». Il est juste de demander un effort de solidarité, provisoire, aux entreprises qui ont engrangé des bénéfices exceptionnels, alors même que l'État a subventionné massivement l'économie dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Ce qui est démagogique, ce sont les impôts différés et non consentis qu'appellera le remboursement de notre dette publique. La proposition, promue par Laurent Lafon, de reporter la suppression de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) répondait aussi à ce problème précis. Nous appelions de nos voeux une large concertation avec le monde de la culture, car remplacer, au pied levé, la CAP par une fraction de TVA ne règle pas la question de l'avenir de l'audiovisuel public. De même, la proposition défendue par notre collègue Michel Canévet, au nom du groupe Union Centriste, sur le financement des frais de carburant répondait à cette philosophie : cibler les aides sur ceux qui en ont le plus besoin, de manière à la fois plus équitable et moins dispendieuse pour la bonne tenue des comptes publics. Prolonger la remise carburant au bénéfice de tous les automobilistes, fussent-ils belges, luxembourgeois ou suisses, pour un coût de l'ordre de 4,5 milliards d'euros, nous paraît peu compatible avec la fin annoncée du « quoi qu'il en coûte ». Au moins avons-nous pu susciter un débat nourri et- il faut le dire -de haute tenue, tout au long de ces deux jours et deux nuits de séance, avec la quasi-certitude et la satisfaction d'y revenir à l'automne prochain, car il y a peu de chances que la dette nous oublie. Néanmoins, nous avons aussi des motifs de satisfaction, bien évidemment, la dotation de soutien en faveur des communes et des groupements les plus fragiles financièrement et les plus affectés par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et par la hausse des prix de l'énergie. Le groupe Union Centriste défendait un « bouclier tarifaire communal ». Il se réjouit d'avoir obtenu, par l'adoption d'un sous-amendement présenté par son président Hervé Marseille, l'extension de la mesure proposée par le rapporteur général Le dispositif final porte à 600 millions d'euros le concours apporté aux collectivités, en y rendant éligibles plus de la moitié des communes. d'hier soir a sauvé cette mesure essentielle pour nos collectivités, et je remercie le rapporteur général, le président de la commission

Félicitons-nous donc de cette compensation à la hauteur des difficultés rencontrées par les collectivités du bloc communal. Pour cette raison déterminante, le groupe Union Centriste adoptera, dans sa grande majorité, ce PLFR. Très bien

aujourd'hui le volet budgétaire. Il s'agissait bien de deux textes distincts, même si d'aucuns ont pu les confondre, les délais d'examen étant, il est vrai, particulièrement resserrés. Je me félicite à mon tour de cet accord en commission mixte paritaire, qui, au-delà de nous éviter encore de longs débats à l'issue incertaine, comme on a pu l'observer hier avec le rejet,

de nos propositions de soutien à la viticulture, durement frappée cette année par la sécheresse et les incendies, et de territorialisation des mesures comme la lutte contre la hausse des prix du carburant. La réforme du financement de l'audiovisuel public est l'un des points importants de ce texte. C'est un sujet déjà ancien, mais auquel il manquait encore l'impulsion politique nécessaire. Nous veillerons néanmoins à ce que l'audiovisuel public continue de bénéficier des financements adaptés à son bon fonctionnement. La renationalisation d'EDF est un autre volet majeur du texte. Je ne reviens pas sur les remarques déjà formulées en première lecture Je note que ce PLFR acte une nouvelle dégradation du solde public, de plus de 15 milliards d'euros. Jusqu'à quand pourra-t-on continuer de financer les déficits accumulés, à l'heure de la remontée des taux d'intérêt ? Espérons que la croissance sera au rendez-vous et nous évitera des hausses d'impôt. Le groupe du RDSE votera donc pour l'adoption de ce PLFR. En conclusion, je tiens à saluer le travail du rapporteur général, la bonne tenue de nos débats et le sérieux de nos discussions, loin de l'ambiance souvent électrique de l'Assemblée nationale. Une chose est sûre : au Sénat, nous n'avons pas de braillards débraillés

Mais l'essentiel de la politique du Gouvernement est matérialisé dans le deuxième texte, ce budget rectificatif, sur lequel nous allons nous prononcer définitivement aujourd'hui. Cette fois, notre vote contre sera sans réserve. En effet, les avancées pour les collectivités locales, mais aussi- je tiens à le souligner -le soutien à l'aide alimentaire, ne masquent pas les graves reculs sociaux, l'injustice profonde et le risque démocratique que contient ce texte, et cela encore plus après la discussion parlementaire qu'avant. tout d'abord. Non seulement il n'y a pas le compte en matière de pouvoir d'achat, car les augmentations prévues restent en dessous de l'inflation, mais, en plus, le détricotage du droit du travail est à l'oeuvre, sans avoir fait l'objet de la moindre concertation sociale. Pour les Français, c'est donc perdant-perdant point de vue de la qualité de vie, faute d'une véritable augmentation des salaires, et perdant en ressources publiques pour financer la protection sociale et les services publics, du fait des mécanismes de désocialisation et de défiscalisation.

voulue par la majorité sénatoriale que d'une mesure exceptionnelle, liée à la période de très forte inflation et censée durer seulement jusqu'en 2023.

Jamais, depuis des décennies, les inégalités de patrimoine n'ont été aussi grandes et, pourtant, vous continuez de refuser tout rééquilibrage fiscal efficace en faisant contribuer les plus aisés, même les multinationales qui tirent un profit incroyable de la situation actuelle des prix de l'énergie : quelque 17 milliards d'euros en un semestre pour TotalEnergies. Vraiment, en cet été 2022, au début d'un nouveau quinquennat, quelle occasion manquée ! ! La taxation des superprofits, beaucoup d'autres pays que la France y viennent, sous une forme ou sous une autre, et même le secrétaire général de l'ONU a plaidé en ce sens avec force, hier. Combien de temps la France continuera-t-elle de ramer à contre-courant ?

il y avait plus urgence à taxer les superprofits des multinationales qu'à remplacer la « redevance télé » par un impôt injuste. Pourtant, vous avez décidé de faire le contraire.

que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. M. le président du Sénat a reçu de reçu de Mme la Première ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.